monsieur le président.

que la restauration concerne également le site dans son ensemble. Outre le parvis, il est demandé qu'une partie des espaces disponibles à l'Hôtel-Dieu soit dédiée à l'accueil des pèlerins, visiteurs et touristes, ainsi qu'à la fonction caritative. En effet, depuis sa construction, la cathédrale a toujours eu une vocation d'accueil humanitaire et caritatif, assurée par l'Hôtel-Dieu voisin. Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, a d'ailleurs proposé, le 18 avril dernier, de mobiliser une partie de l'établissement pour permettre la continuité de l'accueil des pèlerins.

de la commission ? Cet amendement vise à permettre aux fondations privées de prélever une partie des sommes qu'elles auront collectées pour l'aménagement d'une partie de l'Hôtel-Dieu.

Seule la Fondation du patrimoine, de par ses statuts, incorpore dans sa collecte une clause informant les donateurs de la possible réaffectation des fonds à d'autres projets patrimoniaux,

comme le prévoit le décret du 11 janvier 2007 pris pour l'application de l'article 17 de la loi organique du 1 août 2001 relative aux lois de finances. Si la Fondation du patrimoine se voit restituer une certaine somme, elle pourra l'utiliser pour ses autres projets patrimoniaux.

préalable. Néanmoins, eu égard à l'importance des sommes qu'ils se sont engagés à verser, je pense que c'est à eux de choisir à quelle cause ils souhaitent que les dons qu'ils ont promis soient versés, sous réserve que le produit de la souscription

D'éventuelles clauses de réaffectation pourront tout à fait être introduites, si nécessaire, dans ces conventions. Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements.

Cet amendement vise à rendre facultatives les conventions entre l'État ou l'établissement public et les fondations ayant recueilli les fonds au titre de la souscription nationale. Le Gouvernement souhaite inscrire dans la loi la possibilité de conclure des conventions avec les fondations reconnues d'utilité publique chargées de la collecte de fonds, ainsi, le cas échéant, qu'avec les grands donateurs qui voudraient donner directement au Trésor public.

nous ne souhaitons pas que certains responsables ou dirigeants de pays peu démocratiques ou dont l'image laisse penser que leur argent a été mal acquis soient autorisés à contribuer à la restauration de la cathédrale

permettant de refuser et de signaler les dons issus de personnes physiques ou morales susceptibles d'être liées à du blanchiment de capitaux ou de l'évasion fiscale. Il ne s'agit évidemment pas d'instaurer des obligations nouvelles, mais de renvoyer aux dispositifs mis en oeuvre par la DGCCRF, Tracfin et la direction générale des finances publiques pour repérer et sanctionner le blanchiment de capitaux et l'évasion fiscale. Au-delà du seul aspect symbolique, il nous semble qu'il n'est jamais inutile de faire preuve de pédagogie en matière de délinquance financière, surtout s'agissant d'un événement qui,

celle-ci, propre à contribuer à rassurer la plus grande partie des donateurs, qui ne souhaitent pas participer à une opération mal sécurisée financièrement. Quel est l'avis de la commission

Sur les 120 000 édifices religieux répertoriés, environ 30 % manquent d'investissements et d'entretien ; 3 500 églises sont en péril, et il faudrait intervenir rapidement sur environ 5 000 édifices pour qu'ils ne tombent pas en ruines. Or les communes sont responsables de la restauration des églises qui leur appartiennent, contrairement aux cathédrales, propriété de l'État. Il paraît donc naturel que la participation de nos collectivités locales à la collecte nationale mise en place

L'article 5 instaure un régime de défiscalisation dérogatoire pour les dons et versements effectués par les particuliers dans le cadre de la souscription nationale. En portant la part défiscalisée de 66 % à 75 %, dans la limite de 1 000 euros, le Gouvernement souhaite encourager les dons. Toutefois, je crains que la façon d'opérer ne soit pas la bonne, dans la mesure où le choix de la réduction d'impôt ne concernera, de fait, que la moitié des Français : ceux qui sont imposables sur le revenu. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste a déposé un amendement tendant à transformer la réduction d'impôt en crédit d'impôt, afin que les dons de tous les Français bénéficient de la même incitation de l'État.

et l'obligation qui en est résultée pour certaines d'annoncer aussi leur renoncement à la défiscalisation. Ce régime dérogatoire pour Notre-Dame de Paris me conduit à soulever un autre point qui me tient à coeur : le financement de l'entretien de l'ensemble de nos monuments historiques. En effet, on peut s'interroger sur la possibilité de faire bénéficier d'autres monuments historiques, moins connus que Notre-Dame de Paris mais parfois dans un état de conservation dramatique, du même régime dérogatoire, afin de favoriser les dons pour leur restauration. Ce questionnement est d'autant plus légitime que, dans le même temps, il a fallu se battre aux côtés de Stéphane Bern au sujet du reversement des taxes perçues par l'État sur le loto du patrimoine, justement fléché vers les monuments en péril,

dans la mesure où ces derniers sont fondés sur un impôt acquitté par environ 43 % de la population. Il s'agit d'une réelle problématique en termes d'équité fiscale. Nous aurions pu apporter utilement des réponses en la matière.

Bien que le diagnostic sur le coût total de la restauration n'ait pas encore été réalisé, les projections portent à croire que les promesses de don et les dons déjà réunis couvriront le chantier. Il ne nous semble donc pas nécessaire de stimuler une dynamique qui existait antérieurement à cette annonce fiscale.

pourtant les moins aisées, ne feraient l'objet d'aucun soutien fiscal. D'autre part, pourquoi d'autres monuments historiques français, parfois en péril et qui ne jouissent pas du même pouvoir d'attraction que la cathédrale Notre-Dame de Paris, ne bénéficieraient pas du même relèvement de taux ?

En outre, peut-être avez-vous entendu, comme moi, dans le moment d'émotion universelle et de générosité exceptionnelle qui a mobilisé les Français, et pas seulement eux, et qui, je l'espère, continuera de les mobiliser, que, s'il était juste de se mobiliser pour de la pierre- je reprends les termes que certains de nos concitoyens ont utilisés -, il fallait en faire autant pour les hommes et pour les femmes. Je pense qu'il faut entendre ce qui s'est exprimé

Le Gouvernement souhaite, par l'article 5 du projet de loi, encourager un élan populaire autour de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette démarche ne peut qu'être encouragée. le recours à la technique de la réduction d'impôt apparaît en l'espèce sous-optimale dans la mesure où plus de la moitié de la population française- 57 % précisément -ne paie pas l'impôt sur le revenu. En ce sens, l'objet du présent amendement est de substituer à cette réduction d'impôt un crédit d'impôt, qui pourrait concerner, par nature, l'intégralité des donateurs, quelle que soit leur situation fiscale. Aux termes des données disponibles à ce jour, ce sont environ 30 000 dons inférieurs à 1 000 euros qui ont été collectés par les différents organismes concernés. Ainsi, le surplus pour les finances de l'État serait modéré. Lors des débats à l'Assemblée nationale, il a été estimé par le Gouvernement qu'une telle démarche engendrerait une dépense publique supplémentaire. Cependant, il convient de rappeler que le dispositif proposé par le Gouvernement crée lui-même une dépense fiscale supplémentaire pour l'État. De plus, le coût des travaux à engager s'élèverait, d'après les premières analyses, à environ 1 milliard d'euros, ce qui entraînera mécaniquement, au titre de la taxation sur la valeur ajoutée, des recettes pour l'État de l'ordre de 200 millions d'euros. L'argument financier opposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale ne semble donc pas pertinent. En outre, lors de l'examen du texte par la commission des finances, il nous a été opposé que cette proposition était de nature à créer un dispositif fiscal d'exception. d'exception. Les auteurs de cet amendement estiment que cet argument n'est en aucun cas recevable dans la mesure où la quasi-intégralité du projet de loi discuté est d'exception. On vient d'en parler : le rapporteur

le plus opportun.

de l'impôt sur le revenu payé par les Français résidant à l'étranger qui ont des revenus en France et qui, à ce titre, paient leurs impôts en France sur leurs revenus français. Permettez-moi de vous donner les chiffres des prélèvements fiscaux pour les Français résidant à l'étranger, en Europe ou en dehors de la zone Union européenne. prélèvement à la source, la CSG et la taxe exceptionnelle sur les revenus français, au-dessous de 27 519 euros par an, le pourcentage de prélèvement est de 27,5 % pour ceux qui résident dans l'Union européenne et de 37,2 % pour ceux qui résident hors Union européenne ; pour ceux dont les revenus français annuels dépassent le

Malgré cela, leur résidence en France n'est pas considérée comme résidence principale, ce qui les prive de tous les avantages liés à la résidence principale en cas de rénovation, de suppression de la taxe d'habitation, etc. Ils ne sont pas couverts par la sécurité sociale, ils paient donc directement leurs propres assurances santé, la scolarité de leurs enfants. Si mon amendement était adopté, les donateurs ne paieraient pas moins au total, mais une partie irait à l'impôt et l'autre serait fléchée vers la rénovation de Notre-Dame de Paris. Au final, le montant payé, comme vient d'ailleurs de le dire M. le ministre, serait supérieur. nature à conforter les Français de l'étranger dans leur souhait d'être considérés comme des Français à part entière, car ils sont étrangers dans le pays dans lequel ils vivent et aimeraient être Français quand ils sont en France.

d'un comité de contrôle, mais aussi le travail de la Cour des comptes et, éventuellement, celui des commissions intéressées, il y a évidemment de quoi s'assurer de la bonne utilisation des fonds et de la transparence de la collecte.

Le Gouvernement partage votre souhait, monsieur Dominati, qu'une attention toute particulière soit portée aux entreprises, et même aux particuliers, qui connaissent des difficultés économiques liées à l'incendie de Notre-Dame

que ce soit la disposition prévoyant un contrôle des commissions des finances des deux assemblées sur la gestion des fonds ... Si cet amendement est adopté, je démissionne ! ... ou celle disposant que l'établissement public doit communiquer des informations sur la consommation effective des fonds qui lui ont été versés, de manière à pouvoir évaluer si des modifications sont intervenues par rapport à leur affectation initiale.

de la provenance et de l'utilisation des fonds issus de la souscription nationale ne reste pas un voeu pieux, nous souhaitons ajouter aux termes de la loi une date limite pour satisfaire à cette première obligation

des dons, de leur provenance et, surtout, de la façon dont ils seront utilisés. La plus grande transparence est de mise, compte tenu du mode de financement retenu pour la restauration de Notre-Dame de Paris. Il convient de s'assurer qu'aucun euro issu de la générosité des donateurs ne pourra servir à autre chose qu'à la restauration de Notre-Dame

cette question. J'ai déjà longuement développé toutes les raisons qui militent en faveur d'un tel aménagement : les dégâts collatéraux causés par la chute de la flèche et ses particules de plomb, la nécessaire mise en place de structures d'accueil des visiteurs et des fidèles, la nécessaire exposition des collections de la cathédrale, de l'état d'avancement des travaux, voire des fouilles préventives. Dans son rapport annuel sur le montant et l'utilisation des fonds de la souscription, l'établissement public pourra également faire figurer la part de financement affectée

qui relèvent de la compétence de l'État. Or le dispositif de l'article 8 associe le diocèse de Paris au conseil d'administration du futur établissement public chargé des travaux de conservation-restauration de Notre-Dame de Paris. J'aimerais, monsieur le ministre, que vous puissiez dissiper mes inquiétudes sur le respect des équilibres des lois de 1905 et de 1907 à l'aune du contenu de la future ordonnance fixant les règles d'organisation et d'administration de l'établissement public. S'agira-t-il d'une association du diocèse de Paris en vue d'une simple consultation pour recueillir les observations qu'il aura à faire sur la restauration de Notre-Dame ? Ou s'agira-t-il de l'associer aux prises de décision concernant la restauration, avec un droit de vote ou même un avis conforme ? Tout précédent doit être évité. Il ne me semble pas souhaitable de confier à l'Église un pouvoir de décision en matière de maîtrise d'ouvrage, raison pour laquelle je vous demande davantage de précisions sur la forme de cette association qui sera fixée ultérieurement

dispose déjà de structures compétentes comme l'Oppic, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, ou le Centre des monuments nationaux, le CMN, établissement public chargé de chantiers importants, tels que celui de l'hôtel de la Marine ou celui du château de Villers-Cotterêts. mesure générerait inutilement et inéluctablement des coûts et des délais supplémentaires. Or, comme vous le savez, monsieur le ministre, nous sommes aussi en tant que en tant que parlementaires responsables des fonds publics. Nous devons y veiller, comme nous devons veiller à l'efficacité de nos actes.

J'ai l'absolue certitude- on pourrait prendre les paris -que la première chose que fera cet établissement public sera de confier la maîtrise d'ouvrage déléguée à l'Oppic,

pour mener à bien le projet. Par ailleurs, ces opérateurs ne sont pas forcément habitués à conduire des chantiers ouverts, ce qui est l'une des volontés exprimées pour le projet de restauration de Notre-Dame- nous en avons longuement parlé -, afin de mettre à profit ce drame pour relancer et promouvoir les métiers du patrimoine. Il y a donc un vrai risque de déstabiliser leur organisation en leur confiant le projet,

mais serait-ce une réponse appropriée au caractère exceptionnel du chantier de Notre-Dame, à la technicité qu'il requiert et surtout à l'urgence de sa réalisation ? En quoi cette solution permettrait-elle de mieux associer l'ensemble des parties prenantes, diocèse et Ville de Paris compris, à la prise de décision concernant le projet ? Comment garantirait-on la consultation des experts par le biais du conseil scientifique dont les députés ont prévu la mise en place ? Il n'a pas été rare par le passé, comme je l'ai également rappelé lors de mon intervention en début de séance, que la réalisation des grands projets soit confiée à un établissement public. Pour illustrer mon propos, j'ai rappelé le cas du Grand Louvre, de la bibliothèque François-Mitterrand ou, plus proche de nous dans le temps, du musée du quai Branly. Il me semble qu'il s'agit d'une garantie de transparence pour la mise en oeuvre du chantier. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé la création d'un établissement public, considérant que c'était

du ministère de la culture plus largement, l'architecte en chef des monuments historiques, ses confrères et consoeurs font un travail remarquable. Il s'agit d'un travail dans l'urgence.

l'argumentation selon laquelle, parce que vous avez besoin de moyens supplémentaires, il faut créer une nouvelle structure. Comme M.

Le scrutin est ouvert.

Votre amendement tend à supprimer plusieurs modifications apportées par la commission au moment de l'élaboration de son texte et destinées à encadrer davantage le fonctionnement de l'établissement public. Si nous n'avons pas souhaité remettre en cause le principe d'un tel établissement public dédié aux travaux de Notre-Dame, nous avons fait en sorte que sa mission ne déborde pas au-delà. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons précisé qu'il s'agirait d'un établissement public à caractère administratif, comme je l'ai indiqué lors de nos débats en commission. Nous avons également

les tours de Notre-Dame, qui seront inexploitables pendant des années. Il me semble donc que le CMN pourrait avoir son mot à dire sur la restauration pour que, demain, ces tours soient plus facilement accessibles au public payant.

Mon ministère exerce une tutelle sur le Centre des monuments nationaux ; il exercera une tutelle sur le futur établissement public qui sera créé. Il aura donc tout loisir d'écouter les équipes du Centre des monuments nationaux.

Le conseil d'administration doit rester limité aux personnes qui sont véritablement parties prenantes du projet. Il serait incohérent de confier le pouvoir de décision aux commerçants, ou aux associations de riverains, à parts égales avec le propriétaire, l'État, ou l'affectataire.

le ministre : le représentant des associations de commerçants n'a pas d'en ce moment. Il souhaite avoir, très rapidement, un contact avec le ministre de la culture.

l'amendement n° 40. L'élan des souscripteurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, et la place prise par cette restauration parmi les préoccupations des Français depuis le 15 avril méritent que l'on mette en place l'organisation la plus efficace possible pour réaliser ce chantier. Cela nécessite aussi que l'on ne précipite aucune des étapes préalables. Dans cette perspective, les interrogations de la représentation nationale sur l'établissement public, l'opportunité de sa création, son statut et les missions dont il sera chargé doivent permettre de préciser l'habilitation demandée par le Gouvernement pour, éventuellement, créer cet établissement public. Cette transparence et cette exemplarité, nous les devons à nos concitoyens en général et aux donateurs en particulier. C'est justement sur ce point que je souhaite intervenir, car la dernière phrase du premier alinéa de cet contraire à ces principes. Depuis plusieurs années, et dès le début du quinquennat actuel, avec les lois ordinaire et organique pour la confiance dans la vie politique, nous avons fait évoluer notre législation afin de moraliser la vie publique et de garantir l'exemplarité de l'État. Il semble anachronique de trouver dans ce texte une disposition qui prévoit de contourner les règles de la fonction publique pour convenir aux caractéristiques d'une personne en particulier. C'est tout le contraire de l'intérêt général ! Cette disposition vise en effet uniquement à assurer que la personne pressentie pourra prendre la tête de cet établissement et recevoir un traitement en conséquence. Sans préjuger des capacités de la personne concernée à remplir cette mission, de telles pratiques vont à l'encontre de l'exemplarité et ne peuvent manquer de susciter, chez nos concitoyens, une impression de favoritisme et de passe-droit. C'est pourquoi, par cet amendement, je propose la suppression de cette phrase.

45 rectifié. Personne ne pense à avoir des réserves à l'égard de la personnalité envisagée, mais permettre des dérogations aux âges limites prévus pour la fonction publique de l'État, c'est ouvrir une brèche pour l'avenir.

vous avancez. Aujourd'hui, on a bien compris que la solution administrative définitive n'est toujours pas arrêtée : vous ne savez pas s'il y aura un établissement public, quelles seraient sa nature et ses attributions, comment il assurerait la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'oeuvre. Nous vous proposons de préciser C'est ensuite que viendra le temps légitime de nommer son président, mais il ne faut pas faire les choses à l'envers. C'est simplement de la bonne pratique administrative

dès lors que l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public permet déjà aux textes réglementaires qui régiront l'établissement à créer de s'écarter de ces règles.

est plus âgé, c'est une erreur. Ce n'est pas l'âge qui compte, mais l'aptitude. Je veux prendre comme simple exemple une figure qui a marqué l'histoire de notre pays, par rapport aux autres présidents

de conduire la main de la personne qui sera chargée de rédiger le décret de composition de ce conseil scientifique, en lui suggérant de façon assez forte de choisir ses membres au sein des corps de la conservation, des architectes des Bâtiments de France et des architectes en chef des

serait bon de les retrouver dans des structures administratives de l'État. J'ai trop connu d'organismes où, malheureusement, la composition du conseil scientifique

À cet effet, plusieurs informations doivent lui être communiquées chaque année concernant l'affectation et la consommation des fonds. J'ajoute que, depuis 2018, en application de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le ministère de la culture a mis en place un collège de déontologie.

Cet amendement vise à préciser que la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, instituée par la loi de 2016, doit être régulièrement informée et consultée sur l'avancement des études et des travaux.

à l'Assemblée nationale et en commission au Sénat, nous souhaitons que ces ordonnances soient ratifiées dans un délai maximum d'un an après la promulgation du

Il nous semble tout d'abord que la mise en place de telles dérogations n'est pas utile si elle ne vise qu'à accélérer les délais de délivrance des autorisations administratives. Les délais prévus par les différents codes sont des plafonds. Les demandes d'autorisation concernant Notre-Dame peuvent parfaitement être traitées de manière prioritaire

sur l'exemplarité du chantier de Notre-Dame, qui sera particulièrement observé, tant en France qu'à l'étranger, du fait de l'émotion suscitée par le sinistre et du financement de la souscription nationale par un grand nombre de donateurs, qu'ils soient français, européens ou au-delà des océans, comme on disait autrefois. Notre législation particulièrement complète et protectrice en matière de préservation du patrimoine a jusqu'ici été mise en avant par les autorités auprès de l'Unesco pour garantir que la valeur universelle exceptionnelle du site « Paris, rives de la Seine » est protégée, même en l'absence de plan de gestion. Suspendre l'application d'un certain nombre de ces différentes dispositions législatives pourrait constituer une menace pour le maintien de l'inscription de ce bien sur la liste du patrimoine mondial, sachant que le plan de gestion n'en est qu'au stade de l'élaboration et qu'il ne devrait pas être adopté avant encore quelques années. Nous considérons enfin que la mise en place de telles dérogations constitue un danger réel pour la crédibilité de notre législation, déjà mise à mal par les dérogations prévues par la loi Élan votée le 23 novembre 2018, comme

L'État ne peut pas se permettre de s'affranchir de ces lois, même pour l'un des chantiers les plus emblématiques du point de vue du patrimoine, sans prendre le risque de leur remise en cause. Les règles en vigueur apportent, me semble-t-il, une sécurité pour le bon déroulement des chantiers et leurs délais d'exécution, tout en offrant des garanties en termes de transparence et d'acceptabilité.

ne peut pas non plus être l'otage de ce Graal politique qui voudrait que l'on imprime sa marque sur le passé ou dans Paris par un geste architectural à chaque nouvelle mandature. L'audace ne peut être considérée comme l'ultime qualité, se plaçant au-dessus de toute obligation et rigueur, dans les procédures architecturales et patrimoniales. La modernité

Je vous le dis tel que je le pense : la culture, ce n'est pas le productivisme ou le stakhanovisme. Sincèrement, je trouve profondément baroque, triste que ce soit vous, monsieur le ministre de la culture, qui portiez ce texte.

propriétaire de l'ancienne cathédrale, peut-elle accepter de continuer à se soumettre aux différents codes si l'État est autorisé à s'en affranchir ? Il est à craindre que l'exemplarité de l'État, s'octroyant des dérogations en matière de règles d'urbanisme, de protection de l'environnement, de préservation du patrimoine et de commande publique, soit mal perçue par les concitoyens à qui il est demandé de se mettre en conformité avec la législation.

éventuelles et, bien sûr, diagnostic -, mais les dérogations possibles ne la garantissent pas. C'est aussi le cas s'agissant des mécanismes d'autorisation de travaux sur les monuments historiques, qui, selon tous les éléments que j'ai pu recueillir, fonctionnent bien. C'est là la principale raison qui nous a conduits à supprimer cet article en commission des dérogations au droit commun en matière de monuments historiques ou, plus généralement, de patrimoine reviendrait à ouvrir une boîte de Pandore. Comment les élus locaux pourront-ils expliquer que ces dispositions, ces contrôles, ces délais sont essentiels à la préservation du patrimoine, si l'on a pu y déroger pour Notre-Dame de Paris ? Cela reviendrait à montrer

Cet article confirme qu'aucune circonstance ne saurait justifier une loi d'exception. Par le passé, des chantiers de grande ampleur, comme celui de la cathédrale de Strasbourg, ont été menés sans s'affranchir des règles. On ne sait toujours pas pourquoi vous avez souhaité que l'État se soustraie aux règles qu'il impose à tous les citoyens.

sourd aux interpellations de tous ceux qu'inquiète votre volonté de passer outre le code du patrimoine, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, le code de la construction et de l'habitation, le code de la commande publique, le code général de la propriété des personnes publiques, au seul motif d'accélérer la restauration pour tenir les délais présidentiels.

qui sont le triomphe du vide, qui réalisent ce rêve de faire entrer la lumière dans une architecture monumentale défiant les lois de la pesanteur. Elles sont l'aboutissement d'un travail qui a magnifié l'anonymat, les bâtisseurs étant inconnus. reprendre les propos de Sylvain Tesson, aucune signature ne s'associe à leur édification, personne n'est à honorer.

qu'aucun nom d'architecte, connu ou pas, ne vienne « griffer » Notre-Dame de Paris. Nous sommes les dépositaires de ce monument, qui n'est pas un musée. Nous devons le transmettre aux générations qui viendront après nous. C'est pourquoi il ne saurait y avoir de dérogations. Notre patrimoine est respecté dans le monde. Nous savons le préserver, et ce depuis longtemps, selon des règles que nous nous sommes imposées. La valeur

des dérogations aussi importantes aux codes du patrimoine, de l'urbanisme, de l'environnement, des marchés publics. Les parlementaires ne peuvent pas accepter d'aller aussi loin en matière de pouvoirs délégués au Gouvernement.

octroyait un blanc-seing au Gouvernement pour déroger par ordonnances, sans contrôle du Parlement, à l'ensemble des dispositions légales en matière de protection du patrimoine et de l'environnement et aux règles régissant les marchés publics, pour procéder aux travaux de rénovation de Notre-Dame. permettait au Gouvernement de décider, quand bon lui semblerait, de la personne habilitée à gérer les fonds issus de la souscription nationale- l'État ou un établissement public restant à créer -, laissant ainsi planer le doute sur l'utilisation effective des deniers publics pour la restauration de la cathédrale.

de n'avoir pu transformer en crédit d'impôt la réduction prévue pour les donateurs, afin que même les plus modestes d'entre eux, non assujettis à l'impôt, bénéficient d'un avantage fiscal.

commission, modifié, l'ensemble du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. Voici quel